La séance est reprise. La parole est à M. Charles Guené, pour une mise au point au sujet d'un vote.

L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 86 du règlement, au scrutin secret suppléant à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences ; la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie nos collègues MM. Loïc Hervé et Daniel Gremillet, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Le juge suppléant à la Cour de justice de la République nouvellement élu sera immédiatement appelé à prêter serment devant le Sénat.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons donc après que l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, que votre assemblée avait rejeté en votant contre l'article d'équilibre à la fin de l'examen de la première partie du texte. Je ne reviendrai pas sur les dispositions du projet de loi que j'avais eu l'occasion de vous présenter lors de l'examen en première lecture. Je soulignerai simplement que ce projet de loi de finances vise à tenir à la fois les engagements pris par le Président de la République en matière de réarmement des ministères régaliens et de préparation de l'avenir- en témoignent les efforts accomplis dans le domaine de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou encore de la transition énergétique

afin que le plan de relance soit le plus efficace possible. L'Assemblée nationale avait adopté un amendement du Gouvernement visant à permettre la mise en oeuvre sur plusieurs années d'un plan d'investissement pour construire des filières économiques plus compétitives. Elle a ainsi préparé l'économie de la France de 2030.

L'Assemblée nationale a principalement adopté quatre dispositions nouvelles. La première concerne la possibilité qui sera donnée au Gouvernement, si cela se révélait nécessaire, de déroger aux recommandations de la commission de régulation de l'énergie en matière de fixation des tarifs de l'électricité à la fin du mois de janvier, de manière que le bouclier tarifaire mis en place en première lecture soit amélioré et nous permette de faire face à une éventuelle hausse des prix plus importante que prévu. Deuxièmement, nous avons proposé à l'Assemblée nationale, qui a adopté cette mesure, d'abonder à hauteur de 150 millions d'euros un fonds de réassurance, donc de garantie, pour les opérateurs de voyages et de tourisme, afin de les accompagner dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Destination France, mais surtout pour faire

l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à faire de l'État le garant en dernier ressort en cas de déficit dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques. La Ville de Paris s'est engagée dans l'aventure des JO comme ville hôte ; elle a remporté cette bataille aux côtés de l'État. Néanmoins, dans la mesure où la dimension des JO dépasse évidemment le rayonnement de la ville, l'État sera présent en tant que financeur, mais aussi en qualité de garant en dernier ressort. C'est là une disposition que l'Assemblée nationale a adoptée il y a quelques jours.

nous vous présentons un projet de loi de finances qui fixe pour l'année 2021 un niveau du déficit prévisionnel à 8,2 %. Si la croissance devait être supérieure à 6,25 %, cela se traduirait mécaniquement par une diminution des déficits ; tout le monde en serait satisfait.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est pas une surprise, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mercredi 1 décembre dernier, n'a évidemment pas pu établir un texte commun sur le projet de budget, compte tenu de nos points de vue irréconciliables. En première lecture, le Sénat avait rejeté le projet de loi de finances en n'adoptant pas la première partie du texte. Pourquoi le rejet du PLF ? Cela s'explique par l'opposition marquée du Sénat à un budget dont les principales caractéristiques, en termes de montants des dépenses, ainsi que de niveaux historiquement élevés de déficit et d'endettement, ne découlent pas uniquement de la crise épidémique, sociale et économique que la France traverse. En effet, ce budget traduit aussi et surtout des choix budgétaires et fiscaux du Gouvernement auxquels nous nous opposons. nous sommes passés d'un budget initialement « incomplet » à un budget « de campagne », qui, à l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, préempte dangereusement les exercices budgétaires futurs. De très nombreuses mesures ont ainsi été adoptées en dépenses et emportent des conséquences pour les années à venir. Je rappellerai, notamment, le plan d'investissement France 2030 de 34 milliards d'euros- excusez du peu ! -ou encore le contrat d'engagement jeune. Mais de nombreuses autres dispositions pourraient être citées : il y en a pour tout le monde, ou presque ! Par ailleurs, parallèlement aux effets de la crise, le Gouvernement ne maîtrise pas les dépenses qui ne relèvent pas de l'urgence ou de la relance. les dépenses primaires des administrations publiques sont supérieures de plus de 60 milliards d'euros par rapport aux engagements pris dans la loi de programmation des finances publiques depuis 2017. Le niveau des dépenses pilotables de l'État marque également l'absence totale d'effort de maîtrise des dépenses par le Gouvernement. Au-delà des discours officiels, nous assistons à une dérive coupable et assumée des comptes publics. Le Gouvernement hypothèque ainsi sérieusement l'avenir et obère les marges de manoeuvre de la prochaine majorité gouvernementale. Nous considérons également que le Gouvernement ne retient pas les leçons du passé, en faisant le choix de ne flécher aucune recette supplémentaire, issue de l'embellie économique, vers le désendettement de la France. Or les niveaux record de déficit et d'endettement ne peuvent qu'être exceptionnels, et les efforts de maîtrise des comptes publics que nous pourrons réaliser aujourd'hui seront les seront les marges de manoeuvre dont nous disposerons demain en cas de nouvelle crise ou de nouvelle vague. Le projet de loi transmis au Sénat à l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale compte désormais 222 articles, dont 8 supprimés et 7 additionnels. Je rappelle que, en première lecture à l'Assemblée nationale, pas moins de 166 articles additionnels ont été introduits par voie d'amendements. Quelles sont les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et sont-elles de nature à modifier la position exprimée par le Sénat ? Au-delà des 36 articles modifiés pour des raisons purement rédactionnelles ou de coordination, 47 articles ont fait l'objet de rectifications de fond, et beaucoup d'entre eux pour des améliorations purement techniques. Chacun pourra retrouver toutes les modifications dans mon rapport de nouvelle lecture. Je mentionnerai cet après-midi uniquement deux points. Cela ne vous surprendra pas, monsieur le ministre, j'aborderai en premier lieu le « bouclier tarifaire » que votre gouvernement a proposé d'introduire

d'un palliatif mis en place en urgence, qui s'ajoute à la multitude de dispositions déjà adoptées : chèque énergie, indemnité inflation, bouclier fiscal pour l'électricité, bouclier tarifaire pour le gaz, La hausse des tarifs réglementés pourrait ainsi atteindre 20 % en février prochain selon les experts, et le fait de contenir cette augmentation à seulement 4 % pourrait coûter jusqu'à 12 milliards d'euros, soit plus que le rendement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, attendu pour 2022, qui se situe à seulement 7,9 milliards d'euros d'euros ! Le Gouvernement décide de mettre en place, en complément du bouclier fiscal, un bouclier tarifaire qui protégerait temporairement les consommateurs en accompagnant les fournisseurs. Toutefois, la hausse sera « récupérée » ou « rattrapée » sur les factures des consommateurs à compter de février 2023 ! Monsieur le ministre, autant vous le dire franchement : je suis très sceptique. Je ne sais pas exactement comment toutes ces mesures de rattrapage, pour le gaz et l'électricité, seront applicables de façon simultanée, sans que les consommateurs se retrouvent de nouveau en difficulté lors du rattrapage et en garantissant la situation des fournisseurs. Cette mesure me paraît aussi aléatoire que dangereuse. En tout état de cause, ces mesures ne font qu'apporter des réponses ponctuelles, sans que le Gouvernement ait été en mesure de proposer une stratégie de moyen ou long terme sur les énergies permettant permettant d'anticiper les tensions, donc les hausses de prix sur des marchés européens, voire internationaux. Ensuite, l'Assemblée nationale a répondu pour partie aux difficultés soulevées par le Sénat s'agissant de plusieurs mesures. en est-il à l'article 3 du projet de loi de finances relatif au champ du crédit d'impôt en faveur des services à la personne. L'Assemblée nationale a en effet exclu les services de téléassistance et visio-assistance de l'exigence d'inclusion dans une offre globale de services, dès lors qu'il s'agit de services permettant la détection d'un accident à domicile, ainsi que son signalement, et qu'ils sont souscrits au profit d'une personne âgée ou handicapée ou atteinte d'une pathologie chronique qui a besoin de ce type de prestations. Si cette disposition répond en partie à nos inquiétudes, elle en soulève une nouvelle, à savoir la complexité de son application, tandis que, actuellement, le crédit d'impôt bénéficie bien plus simplement aux utilisateurs de tels services. Au total, à l'issue de cette nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le déficit budgétaire est estimé à 153,8 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport à la prévision qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette évolution s'explique surtout par une augmentation de près de 1 milliard d'euros des recettes fiscales nettes et des recettes non fiscales. Le plafond de dépenses du budget général a, quant à lui, été rehaussé à hauteur de 300 millions d'euros et celui des dépenses des comptes spéciaux de 200 millions d'euros. Le besoin de financement de l'État pour 2022 s'établit donc à 297,6 milliards d'euros, contre 302,5 milliards d'euros dans le projet de loi de finances adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Outre la diminution du déficit budgétaire, cette réduction s'explique par la baisse du montant estimé au titre de l'amortissement de la dette à moyen et long termes. la nouvelle lecture réalisée par l'Assemblée nationale, même si elle permet de répondre à certains défauts techniques des dispositions votées en première lecture, ne modifie pas vraiment pas vraiment les grands équilibres et les orientations du budget pour 2022, les améliorations constatées restant mineures et principalement liées à la hausse des recettes. raison pour laquelle la commission des finances propose de confirmer la position du Sénat et de rejeter ce texte par l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable. Je salue notre

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après un examen tronqué du budget en première lecture,

Au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je veux dire de nouveau que nous regrettons le choix de la majorité sénatoriale d'avoir refusé d'examiner mission par mission les dépenses de l'État. Cette posture a privé notre assemblée de l'une de ses missions essentielles, et le manque de respect du Gouvernement pour le Parlement, qui est bien réel, ne saurait à lui seul la justifier.

Républicains, que vous aviez tant de propositions à faire ! Si j'en crois le programme de votre candidate Valérie Pécresse, vous souhaitez réaliser 76 milliards d'euros d'économies d'ici à 2027, diminuer encore davantage les impôts de production, dans une forme de surenchère avec le Gouvernement, et supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Pourquoi ne pas avoir saisi l'occasion de ce dernier budget avant la présidentielle pour illustrer votre programme ? Vous auriez pu ainsi commencer à nous préciser quels postes vous comptez supprimer et dans quels ministères : l'éducation nationale, les forces de l'ordre, nos armées, la présence de l'État dans les territoires ? Nous aurions pu voir

ce dernier budget du quinquennat, qui met fin brutalement au « quoi qu'il en coûte » et qui renoue avec la politique libérale menée depuis 2017, n'aura de conséquences bénéfiques suffisantes ni sur le pouvoir d'achat ni sur l'investissement et la préparation de l'avenir. S'il restait encore le moindre doute chez quelqu'un à gauche, ce dernier budget est celui des dernières illusions perdues. Illusion perdue de la justice sociale, avec une explosion des inégalités de revenus, mais aussi de patrimoine dans le monde entier après cette crise, plus particulièrement dans notre pays, sans que cela semble émouvoir quelque membre que ce soit du Gouvernement ou de la majorité parlementaire. Illusion perdue de la théorie du ruissellement : il n'y a plus aujourd'hui aucun économiste pour donner crédit à cette théorie selon laquelle la politique de l'offre viendrait améliorer la croissance et le sort de l'ensemble de la population, en particulier les plus modestes. Illusion perdue du volontarisme écologique, avec un budget consacré à la transition écologique bien insuffisant et un refus répété de conditionner, écologiquement comme socialement, les aides aux entreprises. entreprises. On se rend compte aujourd'hui que ces aides sont mal calibrées et mal ciblées dans notre pays. Illusion perdue du pouvoir d'achat. Et les dispositions adoptées dans la loi de finances rectificative cet automne ou dans ce projet de loi de finances aujourd'hui, même augmentées de la disposition du nouveau bouclier tarifaire sur l'électricité pour 2022, que vous avez improvisée en vue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ne sont pas à la hauteur des besoins. Les revendications sociales couvent dans notre pays, de manière tout à fait légitime. Illusion perdue, enfin, pour la jeunesse, qui aura été la sacrifiée de cette crise. Même le Président de la République l'a reconnu, sans pour autant en tirer les conséquences en termes de mesures prises dans ce budget, puisque nous aurons finalement, en guise de revenu d'engagement, des contrats d'engagement au compte-gouttes, et puis c'est tout. Finalement, pour résumer, les choix budgétaires constants arrêtés depuis 2017 et qui s'inscrivent de nouveau dans ce dernier budget, malgré la parenthèse du « quoi qu'il en coûte », conduisent en même temps à l'injustice fiscale, à l'insuffisance de la relance et au retard de la transition écologique, tout en conservant un déficit budgétaire élevé- à hauteur de 5 %, avez-vous dit, monsieur le ministre -, mais qui reste bien hypothétique pour l'année 2022. C'est pourquoi notre groupe, regrettant toujours de n'avoir pu discuter, mission après mission, des dépenses de ce projet de loi de finances, votera évidemment sans hésiter contre le projet de loi de finances

Avec 8 % de chômage au quatrième trimestre, la France a atteint sa meilleure performance depuis près de quinze ans, au lendemain d'une crise majeure. Dans ce projet de loi de finances, le Gouvernement nous invite à progresser sur cette voie, avec la poursuite du plan de relance, mais aussi en faveur des investissements d'avenir et des ambitions que porte le plan France 2030 sortir de la crise et regarder vers l'avant ; être présent auprès de chacun, quoi qu'il arrive, mais aussi poursuivre la réindustrialisation de la France ; baisser les impôts tout en contenant le déficit et la dette publics, ... Parlons-en ! ... protéger et accompagner 13 millions de salariés et plus de 2 millions de TPE-PME. Le « quoi qu'il en coûte », tant décrié par les oppositions, a été salutaire pour nos emplois, nos entreprises et notre pouvoir d'achat, dans l'Hexagone comme dans les outremers. d'alléger le fardeau du coût de la vie ; de tenir les engagements pris, comme la suppression de la taxe d'habitation, tout en compensant les recettes des collectivités locales ; de déployer rapidement un bouclier tarifaire contre la hausse des prix du gaz et de l'électricité ; enfin, de prévoir des aides exceptionnelles contre l'inflation pour les foyers les plus modestes, ainsi protégés par une expression de solidarité forte et novatrice. Ce PLF permet de réengager l'État sur ses missions premières- plus de protection, plus de sécurité, plus de justice -, de réarmer les missions régaliennes, avec 1,7 milliard d'euros de crédits de plus pour nos armées,

plan SMA 2025+. Les sujets ne manquent pas. Il y a tant à dire sans doute, tant à débattre assurément, mais surtout à voter, parce que c'est notre rôle. Malheureusement, notre noble représentation a préféré rejeter à une très large majorité l'article d'équilibre et arrêter net l'examen du PLF. chers collègues, je vous le demande : que répondre lorsque les pourfendeurs du Sénat nous diront que notre chambre ne sert à rien ? Le projet de loi de finances sera adopté sans que nous l'ayons amendé ou même sans que nous ayons débattu de ce texte en séance publique. On parle dans certains rangs de « tradition de fin de quinquennat » ... Nous avons des À l'heure où nous prenons la présidence du Conseil de l'Union européenne, à l'heure où les Antilles connaissent une crise forte, à l'heure où de nombreux villages et foyers français ont été submergés par les eaux et la neige, à l'heure où la Nouvelle-Calédonie a choisi la France, ... À l'heure de la campagne électorale ! ... le Sénat décide de prendre des vacances budgétaires, pour mieux se consacrer à l'invective et aux jeux de couloirs Comment dire aux Français et aux élus locaux que nous n'avons pas voulu débattre des moyens consacrés au renforcement des services publics dans les territoires, des maisons France Services, des maisons de santé, de la réduction de la fracture numérique,

finalement, l'examen du projet de loi de finances pour 2022 aura connu une procédure habituelle. J'entends par là que nos débats auront, malgré tout, suivi quelques figures imposées. La première, c'est bien évidemment la traditionnelle motion tendant à opposer la question préalable, déposée par nos collègues communistes. Ils avaient pourtant fait savoir, par voie de presse, qu'ils ne comptaient pas voter la motion que le groupe majoritaire envisageait cette année de déposer. Mais, après que Les Républicains se sont ravisés, ils ont pris leurs responsabilités et déposé leur propre motion. Je tiens ici à saluer leur constance, qui n'a rien à envier à celle de Sisyphe. La seconde figure imposée, à laquelle nous n'échapperons pas non plus cette année, c'est la motion tendant à opposer la question préalable avant la deuxième lecture. Celle-là, comme le veut la tradition, est déposée par la commission, après l'échec de la commission mixte paritaire. On dit souvent qu'il est bon que les traditions ne se perdent pas. En l'occurrence, permettez-moi d'en douter. Car ces deux figures obligées montrent, au fond, que le Sénat est une chambre d'opposition politique, alors qu'elle doit être une assemblée constructive au service de nos territoires. Les élus locaux se moquent bien de savoir si nous rejetons le budget du Gouvernement. Ils veulent savoir comment nous choisissons de les défendre et de les représenter, de façon concrète, par les mesures que nous portons et par les arbitrages que nous prenons.

Ce plan se structure autour de dix objectifs ambitieux pour les investissements publics. Je pense que nous sommes tous convaincus ici qu'il faut donner à la puissance publique les moyens de soutenir et d'accélérer les grandes transitions du siècle. faut nous assurer que la transition climatique ne sera pas une variable d'ajustement budgétaire, mais sera programmée sur le temps long. Ainsi, quelque 30 milliards d'euros ont été inscrits dans le marbre de la loi. C'est énorme, mais la réussite d'un plan ne réside pas dans les crédits mobilisés ; en cela, je rejoins le rapporteur général. Il faut que l'argent soit utilement fléché dans nos territoires, de façon opérationnelle, en lien avec nos collectivités locales et le tissu économique. Il faut que ce plan retisse la fibre de nos territoires. Nous avions là un rôle important à jouer. Pourtant, la majorité d'entre nous a volontairement renoncé au débat, tandis que les élus locaux, nos mandants, attendaient que nous nous fassions leur porte-voix. J'aurais aimé, aussi, formuler des propositions sur les outils que nous comptions mettre en place pour mobiliser l'épargne des Français. Celle-ci n'est pas dans son état le plus dynamique sur les livrets, alors que les besoins de financement des transitions écologique et numérique sont massifs. J'aurais également aimé vous faire des propositions concrètes pour optimiser l'immobilier universitaire, un sujet sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler au nom de la commission des finances. Enfin, j'aurais évidemment souhaité que nous puissions formuler des propositions pour renforcer l'efficacité de la justice, pour mieux décarboner notre économie, ou encore pour renforcer la sécurité des Français. Bref, cette deuxième partie aurait été l'occasion pour nous de faire valoir nos positions, non pas sur des considérations d'ordre général, mais sur des questions bien précises. Je regrette sincèrement que le Sénat se soit ainsi privé de l'occasion d'examiner le budget dans sa totalité. Notre groupe, qui tient

Cette décision exceptionnelle a été prise pour alerter l'opinion sur la gravité de la situation de nos finances publiques. Celle-ci a été, bien sûr, fortement aggravée par la crise économique liée à la crise sanitaire, qui a nécessité l'adoption de nombreuses mesures coûteuses pour faire face à l'urgence et sauvegarder, puis relancer, notre économie. Nous ne contestons pas la nécessité de ces dépenses. Nous les avons même soutenues, en adoptant tous les projets de loi de finances rectificative qui les ont mises en oeuvre. En revanche, la situation extrêmement dégradée de nos finances publiques- publiques- je le rappelle, nous nous situons en queue de peloton de l'Union européenne pour quasiment tous les indicateurs -résulte également de la gestion de nos finances en dehors de la crise. Comme l'a rappelé notre rapporteur général à plusieurs reprises, les dépenses ordinaires, c'est-à-dire non liées à l'urgence ou à la relance, ont dérivé de 60 milliards d'euros durant ce quinquennat par rapport à l'objectif que s'était fixé Emmanuel Macron au début de son mandat, dans la loi de programmation des finances publiques. Monsieur le ministre, vous avez annoncé à plusieurs reprises la fin du « quoi qu'il en coûte ». Dès janvier 2021, il y a presque un an, vous expliquiez : « Le : « Le niveau de dépenses que nous connaissons aujourd'hui n'est pas soutenable dans le temps. » Pourtant- c'est ce que nous avons voulu dénoncer par notre vote négatif, en refusant d'examiner le volet dépenses du projet de loi de finances -, depuis trois mois, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre n'ont cessé d'annoncer de nouvelles dépenses sans aucun lien avec la crise, une succession de chèques en bois qui a fait exploser le compteur. La plupart de ces mesures ont été intégrées au fil de la discussion budgétaire, sans étude d'impact- faut-il le rappeler ? -, ce qui, au regard des montants en jeu, soit plusieurs dizaines de milliards d'euros, est du jamais vu Nous pouvons vous détailler l'objet de ces annonces, mais vous les connaissez, et la liste a été reprise dans la presse. Je tiens cependant à en rappeler les montants, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre ce que signifie la fin du « quoi qu'il en coûte » ... Le 2 septembre, ce fut une

mes chers collègues, pour cette énumération fastidieuse, mais elle me semblait nécessaire pour mettre en lumière, de manière manifeste, la contradiction avec la prétendue fin du « quoi qu'il en coûte » ! À cette liste, je pourrais ajouter l'annonce, il y a une semaine, de 350 millions d'euros de prime de Noël.

25 milliards d'euros en trois mois, c'est entre 200 et 300 millions d'euros promis en moyenne chaque jour ! Jamais un Noël n'aura été aussi faste ! Manifestement, le père Noël Macron confond le calendrier de l'Avent avec le calendrier électoral. Excellent

Les enfants, en grandissant, apprennent que ce sont les parents qui paient leurs cadeaux. Avec le père Noël Macron, la réalité est bien pire encore : les cadeaux sont pour les parents et sont payés avec la tirelire de leurs enfants et petits-enfants ce n'est pas le père Noël, c'est le père Fouettard ! Il faudrait savoir ! Au regard de cette situation et de notre position en première lecture, il est inutile de refaire le débat et de réexaminer le budget, puisque les mêmes causes auront les mêmes conséquences.

les décisions de justice pleuvent et se ressemblent ! Le 19 novembre 2020, le Conseil d'État, saisi par l'Affaire du siècle et la mairie de Grande-Synthe, observait que la baisse des objectifs de diminution des gaz à effet de serre pour la période 2019-2023 remettait en cause la possibilité pour la France de respecter l'accord de Paris

quinquennat : la place des personnes en situation de handicap dans notre société. On cite souvent le problème de la conjugalisation de l'AAH, qui met sous tutelle toutes les personnes handicapées, mais on pourrait aussi évoquer le budget de l'éducation nationale. À travers toute la France,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen du dernier budget du quinquennat entérine une crise démocratique majeure, qui ne peut être circonscrite aux seules assemblées. La recomposition du rôle du Parlement dans la procédure budgétaire alimente la défiance citoyenne à l'égard de la démocratie. Si des facteurs institutionnels en sont la cause, le problème qu'ils posent ne doit pas dédouaner les majorités La République En Marche et Les Républicains. L'inversion du calendrier électoral déresponsabilise les députés au profit d'un présidentialisme exacerbé. La société civile s'est d'ailleurs détournée des travaux budgétaires. ont les yeux rivés sur le casting présidentiel, beaucoup d'autres sont en grève politique. Tous sont préoccupés par la santé. Citoyens, associations, ONG, syndicats ont bien reçu le message : ce débat est une mascarade.

Le désendettement, priorité ultime pour certains, passerait exclusivement par la réduction des dépenses publiques. Il n'est jamais question d'une réduction des niches fiscales et d'un accroissement de la contribution de quelques privilégiés ! Rétablir

à la réalité, faite, elle, d'injustices et d'inégalités. Le Gouvernement consent peu pour les plus précaires et même pour le plus grand nombre. Lorsqu'il daigne écouter le groupe communiste- ça lui est arrivé ! -,

... On use d'une parade hypocrite : la prétendue menace d'une censure constitutionnelle permet de faire accepter un calendrier de hausse des prix de l'électricité. nous avons un amendement tout prêt, qui, s'il était adopté, permettrait de faire peser cette augmentation sur les fournisseurs d'électricité, qui réalisent des profits exceptionnels grâce à l'envolée de plus de 25 % des tarifs annoncés sur l'année. Nous constatons une forme de lassitude des Français, qui n'attendent plus rien de ce gouvernement. Marcel Proust abonderait par ces mots : « Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. » Le dernier budget du quinquennat est à l'image des précédents

en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2022 s'accompagne d'une impression de déjà-vu. Après le rejet de la première partie du projet de loi de

Nous l'avons dit et nous vous le redisons aujourd'hui : les membres du groupe Union Centriste auraient souhaité procéder à une première lecture pleine et entière de cet ultime projet de budget du quinquennat, non pour donner un blanc-seing au Gouvernement, mais précisément pour tenter d'y apporter des améliorations, dans un esprit de responsabilité budgétaire. Nous devons, hélas, constater que le creusement de la dépense et du déficit est au coeur de ce budget. Qui paiera demain pour rembourser cette dette abyssale ? Les Français, et notamment les plus jeunes

De la même façon, nous avons souligné l'effort financier en faveur des collectivités territoriales, à l'instar de la prolongation en 2022 du dispositif de soutien aux équipements publics locaux et de la dotation C'est donc dans un esprit de sagesse que nous avions déposé un certain nombre d'amendements visant tout à la fois à permettre de meilleures rentrées fiscales et de moindres dépenses budgétaires. Nous avions, par exemple, proposé de transformer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintroduire dans l'assiette fiscale de l'IFI le patrimoine polluant dit « luxueux Nous avions également proposé un renforcement de la lutte contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes, afin d'endiguer ce phénomène préjudiciable pour nos finances publiques autant que pour le civisme fiscal. Sous l'impulsion de nos collègues Sylvie Vermeillet et Bernard Delcros, notre groupe avait par ailleurs dégagé des pistes d'économies, sur lesquelles il eût été à l'écoute de tous les avis constructifs si nous avions débattu du budget jusqu'au bout.

si le Gouvernement surfe désormais sur l'idée du « quoi qu'il arrive », nous devons nous soucier aussi de l'avenir de nos comptes publics. Voulons-nous réellement laisser aux futures générations un désordre budgétaire structurel, marqué par une effervescence dépensière avant chaque élection présidentielle ? ? Une partie de la hausse des dépenses publiques ordinaires dans ce projet de loi de finances n'est pas sans rappeler le dernier budget de la mandature de François Hollande. Je m'inquiète légitimement de la récurrence de cette pratique. Une règle d'or pourrait être instituée afin que nos comptes, déjà fortement dégradés, ne soient pas tous les cinq ans

le groupe Union Centriste réaffirme l'impérieuse nécessité d'engager un assainissement des comptes publics, qui ne soit pas incompatible avec la croissance économique et le bon fonctionnement des services publics. L'État peut légitimement s'endetter, mais uniquement dans le cadre d'une relance économique.

Au nom du groupe du RDSE, le président Requier a expliqué les raisons de notre désaccord avec le vote majoritaire du Sénat lors de l'examen du dernier budget du quinquennat, lequel est aussi le plus coûteux

le groupe du RDSE a voté en faveur de la première partie du projet de loi de finances afin d'inscrire les amendements dans la loi et de poursuivre la discussion budgétaire.

De plus, l'interruption de la discussion budgétaire en première lecture a réduit à néant nos espoirs d'améliorer le projet de loi de finances. Les amendements adoptés ici sont restés lettre morte. Je pense à celui de notre collègue Éric Gold

Monsieur le ministre, vous revendiquez un budget « sur mesure », un budget du « quoi qu'il arrive », qui remplace le « quoi qu'il en coûte ». L'une de ses principales mesures vise à limiter l'effet de la hausse des prix de l'énergie sur le pouvoir d'achat des Français. la possibilité de bloquer unilatéralement la hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité et le versement d'une prime de 100 euros. Avec ce budget, l'endettement de la France va se maintenir bien au-delà des 110 % du PIB en 2022.

de la commission des finances de la qualité de nos échanges. Je ne voudrais pas les compromettre en disant que les heures passées ensemble au banc ont forgé des liens de sympathie et d'amitié, je ne le dirai donc pas ... À travers eux, je souhaite remercier les sénatrices et les sénateurs qui ont participé au débat, plus particulièrement les responsables des différents groupes, en tout cas

séance est suspendue.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

de Belenet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est proclamé juge suppléant à la Cour de justice de la République. de la République, va être appelé à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs On est de son enfance comme on est d'un pays. » Ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry résonnent en chacun de nous : l'enfance est ce pays qui nous a vus naître et grandir, qui nous forge et nous construit, cette terre empreinte de nos joies et de nos souffrances, qui ne nous quittera plus jamais totalement et sera le compagnon de nos vieux jours. Elle est ce « sol sur lequel nous marcherons toute notre vie », nous dit la poète Lya Luft. Mais ces mots ne révèlent-ils pas autre chose, ne laissent-ils pas entendre, aussi, qu'un pays se définit par le sort qu'il réserve à son enfance, à ses enfants ? Le texte que nous examinons aujourd'hui n'aborde pas toutes les facettes de l'enfance dans notre pays : il se concentre sur l'enfance protégée, sur ce que l'on appelle communément la protection de l'enfance, dont l'incarnation institutionnelle est l'aide sociale à l'enfance (ASE). Ce texte est important pour plusieurs raisons.

notre système de protection de l'enfance s'est progressivement renforcé. Il épouse autant qu'il traduit la perception que la société a de la famille, des liens qui régissent cette dernière, de la place et du statut que l'enfant occupe en son sein, et donc en réalité au sein de la société tout entière. D'abord D'abord objet d'attention, l'enfant a progressivement conquis son autonomie pour sortir de son statut d'adulte en devenir au sein d'une famille, laquelle a évolué en même temps que la société autour d'elle.

prendre ses responsabilités, tout simplement parce que la vie d'un enfant protégé, comme celle de tout enfant, n'a pas à pâtir des subtilités de notre organisation administrative et politique.

L'État a également investi massivement dans la pédopsychiatrie pour rattraper vingt ans d'abandon de cette discipline, des enfants et des professionnels qui s'en occupent. L'État a mobilisé, de façon prioritaire pour les enfants sortants de l'aide sociale à l'enfance, l'ensemble des dispositifs de droit commun afin de les accompagner progressivement vers l'autonomie.

Cette vision part de l'enfant et de ses besoins fondamentaux, et non des structures, de notre organisation ou des compétences des uns ou des autres. Elle reconnaît le besoin de protection de l'enfant en tant qu'être intrinsèquement fragile, en tant que sujet de droit, afin de garantir son développement et son épanouissement. Cette protection n'est pas forcément institutionnelle, mais quand elle l'est, elle doit être sans faille. Elle doit garantir à l'enfant sa sécurité affective, physique et matérielle, ce « méta-besoin » sans lequel rien d'autre ne peut se construire, sans lequel aucun autre besoin ne peut être satisfait, sans lequel son accès à l'autonomie pleine et entière n'est pas possible, sans lequel ce sol sur lequel on marche toute sa vie cette protection ne peut pas être exclusivement institutionnelle. Méfions-nous au contraire d'une approche trop mécaniquement et systématiquement institutionnelle, qui ne donnerait aux enfants que la perspective d'être protégés par des murs. Ce ne sont pas les murs qui protègent : parfois même, c'est quand les murs sont trop épais ou trop hauts que le danger rôde et revient. Ce sont non pas les murs qui vous protègent, mais les gens qui vous entourent et qui prennent soin de vous, les liens qui vous sécurisent sur le plan physique et affectif.

La vision politique de la protection de l'enfance que je porte depuis trois ans consiste ainsi à renforcer, à mobiliser davantage et à sécuriser les trois cercles de protection entourant l'enfant, à sortir d'une approche parfois encore trop institutionnelle dans notre pays, comme cela a pu être le cas pour d'autres fragilités, comme le handicap ou la dépendance.

Bien qu'investis de l'autorité parentale, tous les parents ne disposent pas forcément de compétences parentales innées, mais en chacun peuvent sommeiller des ressources que nous nous devons d'identifier, de stimuler et d'étayer pour que l'enfant

Il n'est pas question de revenir à une vision trop familialiste ou parentaliste de la protection de l'enfance. C'est bien l'intérêt supérieur de l'enfant qui constitue la boussole unique guidant chacune des décisions prises en responsabilité par le juge, par le travailleur social, par le personnel de santé,

d'ailleurs Corinne Imbert - facilite l'adoption par les familles d'accueil en les dispensant de la procédure classique, quand la tata est devenue famille à part entière. Alors que la stratégie de prévention et de protection de l'enfance prévoit déjà le financement par l'État de 10 000 parrains

ces deux premiers cercles de protection ne suffisent plus pour répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant et lui garantir la sécurité affective et matérielle nécessaire à son épanouissement. Se met alors en place, par voie administrative ou judiciaire - les deux voies étant parfois complémentaires -, tout notre système de protection institutionnelle

C'est ce qui conduit également le Gouvernement à organiser à la mi-janvier une conférence sur les métiers du social et du médico-social, pour répondre plus largement aux attentes des travailleurs sociaux. Ainsi, quand l'institution recouvre les enfants de son voile protecteur, elle ne peut qu'être bienveillante, sécurisante, rassurante et enveloppante. Elle doit leur permettre de mener la vie d'un enfant comme les autres, ni plus ni moins, ce qui est à la fois très simple et extrêmement compliqué partir à l'étranger avec les copains de sa classe, ne plus être séparé de ses frères et soeurs et vivre à leurs côtés, par exemple. Cette institution ne peut pas laisser la moindre place à une quelconque forme de violence de la part des adultes. Elle doit aussi parfois veiller à protéger les enfants des autres enfants et parfois même les enfants contre eux-mêmes. Pis, on ne peut tolérer que l'institution engendre elle-même de la maltraitance et de la violence, en imposant par exemple de multiples ruptures à des enfants déjà marqués par une séparation souvent traumatisante dans leur jeune existence.

départements, les associations et l'État, chacun à son niveau, afin que la sécurité physique des enfants soit garantie, notamment en instituant un référent extérieur auquel les enfants pourront s'adresser en cas de violence subie ou constatée. En parallèle, dans la continuité des travaux déjà effectués par le Conseil national de la protection de l'enfance, nous travaillons avec les acteurs sur la fixation de normes et de taux d'encadrement afin que les décrets puissent être publiés avant la fin du quinquennat.

L'Assemblée nationale a adopté le principe de cette interdiction, en encadrant strictement les exceptions : le rapporteur Bernard Bonne vous proposera un dispositif sensiblement différent, auquel adhère le Gouvernement. J'évoquais à l'instant les ruptures encore trop nombreuses que vivent un certain nombre d'enfants au sein de notre système institutionnel de protection de l'enfance. Il en est une qui, lorsqu'elle se produit, est particulièrement dramatique pour l'enfant, parce qu'elle met à bas tout l'investissement consenti auparavant : c'est la rupture que connaissent certains jeunes en sortant du dispositif de l'aide sociale à l'enfance.

accompagnement, bourse étudiante, logement étudiant, logement social. L'Assemblée nationale a encore renforcé l'accompagnement des jeunes majeurs, en votant par exemple l'accès automatique à la garantie jeunes pour ces jeunes. En commission, le rapporteur Bonne a formellement consacré un droit au retour pour tout jeune de l'aide sociale à l'enfance qui rencontrerait des difficultés qu'il n'avait peut-être pas anticipées. Je vous propose aujourd'hui d'aller plus loin encore, avec un objectif simple en finir avec le couperet des 18 ans, qui fait trop souvent office d'épée de Damoclès pour les jeunes protégés. Il faut, d'une part, systématiser l'accompagnement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance de 18 à 21 ans d'autre part, rendre obligatoire la mise en place pour chaque jeune d'un projet pour l'autonomie, qui prolonge et complète le projet pour l'enfant, qui soit adapté à la situation, aux besoins et aux envies de chacun. Ce projet pour l'autonomie reposera sur trois volets.

et de leurs responsabilités. L'État sera aux côtés des départements puisque, dès l'adoption de la loi, État et départements travailleront ensemble sur les détails précis de l'accompagnement financier de ces derniers.

Bonne et de l'ensemble des sénatrices et sénateurs ayant contribué à ce texte, notamment sur la question de la gouvernance locale, qui va constituer, j'en suis convaincu, un apport majeur du Sénat. Ce processus a aussi pleinement associé les enfants eux-mêmes et je conclurai sur ce point. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance présentée en octobre 2019, j'avais souhaité accorder une place importante à la question de la parole des enfants protégés, afin que ceux-ci puissent être pleinement acteurs de leur parcours et être associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques qui les concernent. Il est temps que le champ de la protection de l'enfance accorde davantage aux enfants les moyens d'agir et de garantir leurs droits. Trop souvent, les enfants protégés manquent d'espaces pour s'exprimer sur leur quotidien, sur les aspects positifs et négatifs de l'environnement dans lequel ils évoluent. Il faut pourtant leur donner la parole pour qu'ils puissent partager leur vision, leur vécu,

par des sénateurs ou par le Gouvernement, à commencer par l'audition systématique de l'enfant par le juge, que je vous proposerai d'adopter à l'article 7 du projet de loi. Le résultat de ces travaux d'enfants ou d'anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance montre d'ailleurs parfaitement que la protection de l'enfance est une question très complexe, qui autorise difficilement les raisonnements simplistes ou les solutions toutes faites. Ce n'est pas ce qui est blanc ou noir qui pose question ; ce sont souvent les nombreuses nuances de gris qui soulèvent le plus de difficultés, interrogent nos pratiques et nous mettent au défi. Méfions-nous d'ailleurs des discours exclusivement négatifs. discours exclusivement négatifs. Racontons aussi les belles histoires de la protection de l'enfance, parce qu'elles sont valorisantes pour l'ensemble des enfants et pour les professionnels qui sont à leurs côtés. ! Nous avons la même boussole que les professionnels, qui, à leur place, dans leur rôle, protègent les enfants au quotidien : cette boussole, c'est bien évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant. Notre responsabilité commune est de les aider et de les guider dans cette tâche, avec l'humilité de ceux qui n'expérimentent pas dans leur quotidien, dans leur conscience et leur chair, la complexité que peut constituer le fait de décider pour un enfant et pour son avenir, pour lui et avec lui. Je suis convaincu qu'avec ce projet de loi, nous oeuvrons tous ensemble en ce sens. La parole

la hausse constante du nombre de mesures d'aide sociale à l'enfance montre l'attention croissante que la société porte à la protection des enfants, dans le contexte d'une libération de la parole et d'une meilleure prise en compte des phénomènes de maltraitance. En 2018, les départements ont ainsi mis en place 355 000 mesures d'aide sociale à l'enfance, pour une dépense de 8,3 milliards d'euros. D'importants progrès ont été réalisés pour améliorer la protection des enfants en danger, en particulier grâce aux lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016. Ces avancées connaissent toutefois une application bien trop inégale selon les territoires. La déjudiciarisation de la protection de l'enfance n'a pas eu lieu, 80 % des placements étant encore ordonnés par le juge. Le projet pour l'enfant n'est pas systématiquement mis en oeuvre et les observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) ont des moyens très variables selon les territoires. Si le département est chef de file, la protection de l'enfance fait intervenir de nombreux acteurs, en particulier l'autorité judiciaire et les services de l'État. Or ces acteurs sont insuffisamment coordonnés et fonctionnent encore trop en silos, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local : nous manquons d'outils efficaces de pilotage et d'évaluation. Le bon fonctionnement de la protection de l'enfance repose ainsi sur la volonté de chaque département et de ses partenaires. De nombreux professionnels et élus se mobilisent, dans des conditions souvent difficiles, pour assurer une prise en charge de qualité des enfants en danger. Pour autant, force est de constater que cette politique publique manque d'efficience, que les prises en charge des mineurs protégés sont plus ou moins satisfaisantes et que l'accent n'est pas assez mis sur la prévention des carences éducatives. Les jeunes sortant de l'ASE rencontrent d'importantes difficultés d'insertion sociale et professionnelle, 70 % d'entre eux n'ayant aucun diplôme, ce qui témoigne d'une forme d'échec de la protection de l'enfance eu égard aux moyens qui

Les principes sont posés par les lois de 2007 et de 2016 ; il s'agit non pas de les réinventer, mais de les appliquer. Dans cette logique, le projet de loi ne porte pas de réforme en profondeur de la protection de l'enfance, mais entend ajuster les modalités d'accompagnement des mineurs, mieux prévenir les risques de maltraitance et unifier la gouvernance nationale. La commission partage ces objectifs. Nous avons travaillé dans la perspective d'apporter d'utiles compléments aux travaux déjà menés tant par le Gouvernement que par nos collègues députés. Nous devons apporter des outils concrets complémentaires à ceux qui existent déjà, afin de coordonner et d'harmoniser les prises en charge, de faciliter les diverses modalités d'accompagnement des enfants et d'améliorer la gouvernance, en particulier à l'échelon local. concerne l'accompagnement et l'accueil des mineurs et des jeunes majeurs protégés, la commission a soutenu les mesures favorisant l'accueil des enfants par un tiers digne de confiance et leur accompagnement par des parrains ou marraines. La commission a ensuite approuvé et enrichi l'article 3 D, qui prévoit des mesures de lutte contre les sorties sèches. Le texte prévoit que la garantie jeunes sera systématiquement proposée aux jeunes de l'ASE éligibles. De même, les jeunes majeurs de moins de 21 ans en difficulté d'insertion sociale devront être pris en charge temporairement par l'ASE. La commission a consacré un droit au retour en s'assurant que l'accompagnement des jeunes majeurs sera possible, y compris s'ils ne bénéficient plus d'une prise en charge. L'accompagnement des jeunes majeurs représente une charge nouvelle pour les départements, alors que le Gouvernement est resté évasif sur la compensation de cette charge par l'État. Aucun crédit n'a été budgétisé dans le projet de loi de finances pour Si les arbitrages précis sur les modalités de calcul ne sont encore pas rendus, des engagements en faveur d'une réelle compensation financière sont attendus. La commission a complété le texte pour mieux encadrer les types de structures accueillant les mineurs et renforcer la lutte contre les maltraitances ou les situations d'enfance en danger. Alors que l'accueil de mineurs à l'hôtel ne constitue en aucun cas une solution, entre 7 500 et 10 000 mineurs protégés y sont hébergés aujourd'hui. Face à cette situation inacceptable, la commission a renforcé les dispositions de l'article 3 afin d'interdire totalement l'accueil à l'hôtel dans un délai de deux ans. La commission a supprimé la création d'un droit de visite des parlementaires dans les établissements de l'ASE, car ce ne sont pas des lieux de privation de liberté. Cette mesure est contre-productive, tant pour la protection des enfants que pour les prérogatives du Parlement. Nous avons précisé le contenu de l'article 4 afin que les contrôles des antécédents judiciaires du personnel et des bénévoles exerçant dans le secteur social s'appuient sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Le référentiel national d'évaluation des informations préoccupantes prévu à l'article 6 permettra d'harmoniser les pratiques et de se conformer aux meilleurs standards scientifiques.

Afin d'améliorer la procédure d'assistance éducative, la commission a approuvé la possibilité de renvoyer une affaire particulièrement complexe devant une formation collégiale, ainsi que celle donnée au juge de désigner un avocat pour l'enfant, en ajoutant que cette désignation pourra être demandée par le président du département. Nous aurons d'ailleurs l'occasion, lors de nos débats, de discuter des modalités de représentation et de prise en compte de la parole de l'enfant. Le texte consacre plusieurs dispositions aux assistants familiaux, dont le déclin démographique pose des difficultés majeures. La commission a soutenu la sécurisation de leur rémunération au niveau du SMIC dès le premier enfant accueilli et le maintien de la rémunération en cas de suspension de l'agrément. Nous avons également complété ces dispositions afin de renforcer la place des assistants familiaux dans l'élaboration et le suivi du projet pour l'enfant. La commission a adopté l'article 11 permettant à l'assistant familial de travailler au-delà de la limite d'âge pour prolonger l'accompagnement d'un enfant. L'article 10 prévoit la création d'une base nationale répertoriant les agréments des assistants familiaux afin que chaque département puisse avoir connaissance des retraits ou des suspensions d'agrément sur l'ensemble du territoire. Saisissant l'opportunité que constitue la création de cet outil, la commission a ajouté à cette base les agréments des assistants maternels. La commission a modifié l'article 12, qui instaure des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection maternelle et infantile en renforçant le rôle des départements dans la définition de ces priorités. Nous avons également maintenu les normes minimales d'activité des PMI et d'effectifs de professionnels de santé s'imposant aux départements, aux côtés des nouveaux objectifs nationaux de santé publique que le texte institue. Il s'agit d'éviter de passer à une logique de résultats sans une garantie minimale sur les moyens accordés à la PMI. En matière de gouvernance, l'article 13 prévoit de regrouper les instances nationales oeuvrant dans le champ de la protection de l'enfance au sein d'un seul groupement d'intérêt public qui aura pour mission d'élaborer des référentiels et de diffuser de bonnes pratiques. Cette réforme devrait permettre de mieux coordonner les acteurs nationaux et d'améliorer la connaissance et l'harmonisation des pratiques professionnelles. Il conviendra toutefois que les acteurs concernés travaillent réellement ensemble en ayant les moyens de le faire, sans quoi ce GIP restera une coquille vide sans réelle valeur ajoutée. La commission a supprimé la mission confiée aux ODPE d'organiser une gouvernance territoriale renforcée, car il n'est pas opportun d'assigner une telle mission à des observatoires qui disposent de moyens très variables. Pour améliorer la gouvernance territoriale, nous avons introduit l'expérimentation, dans les départements volontaires, d'un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du département et le préfet. Cette instance permettra de réunir l'ensemble des acteurs locaux de la protection de l'enfance pour coordonner leurs actions, définir des orientations communes et traiter de situations individuelles complexes. Elle contribuera ainsi à une meilleure articulation des acteurs intervenant auprès des enfants, afin de leur garantir une prise en charge transversale et sans rupture de parcours. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés (MNA), nous avons regretté que le texte n'organise pas le transfert à l'État de l'exercice et du financement de la compétence de mise à l'abri, d'évaluation de la minorité et d'isolement des personnes se déclarant MNA. La commission a toutefois soutenu les dispositions de l'article 14, qui prévoit une répartition plus juste des MNA sur le territoire. Elle a complété l'article 14 afin d'étendre l'interdiction faite aux départements de procéder à des réévaluations de la minorité à tous les MNA reconnus comme tels par l'autorité judiciaire.

Ce texte comporte des mesures utiles pour faciliter et harmoniser les pratiques professionnelles sur le terrain, afin de mieux prévenir les situations de danger et de protéger les enfants. Ces mesures auront toutefois un coût pour les collectivités. Si l'on veut s'assurer de leur mise en oeuvre effective, il conviendra que l'État accompagne financièrement les départements. C'est la condition d'une véritable application de la loi et d'une protection efficace des enfants sur tout le territoire de la République. La parole

lesquels : des enfants au parcours de vie souvent difficile, voire chaotique, qui doivent être protégés et accompagnés. Le sort de ces enfants, qui se considèrent bien souvent comme les « enfants de personne », est aujourd'hui au coeur de nos débats. Ma satisfaction, ensuite, car ce texte comporte, monsieur le secrétaire d'État, de belles avancées pour améliorer le quotidien et l'accompagnement des enfants sous protection. J'y reviendrai. Malgré les avancées majeures que les lois de 2007 et de 2016 ont consacrées, de nombreux dysfonctionnements subsistent et nécessitent un renforcement de notre système de protection de l'enfance. Ce projet de loi prévoit ainsi de changer le regard que la société porte sur les enfants pris en charge par l'ASE, l'objectif étant de garantir leurs droits. Il s'inscrit ainsi dans la stratégie globale proposée au Gouvernement par la commission des 1 000 premiers jours, présidée par Boris Cyrulnik et qui a fait l'objet d'une large concertation. Ce texte, je le disais, comporte de belles avancées. Je pense ainsi à l'accueil prioritaire des fratries dans un même lieu, car nous ne pouvons tolérer que soient séparés des frères et soeurs qui partagent des liens affectifs et une histoire commune.

Je pense également au renforcement du contrôle du personnel exerçant dans le secteur social et médico-social, mais aussi à celui de la prévention et de la lutte contre la maltraitance, ainsi qu'à la création d'un référentiel national d'évaluation des situations de danger

Je pense enfin aux dispositions relatives au pilotage de la politique de prévention et de protection de l'enfance, ainsi qu'aux mesures qui permettront de mieux protéger les mineurs non accompagnés, dans la continuité des propositions que Laurent Burgoa, Hussein Bourgi, Henri Leroy La protection des enfants doit nous rassembler au-delà des clivages qui existent au sein de cet hémicycle, car nous, parlementaires, sommes aussi des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes et peut-être même d'anciens enfants placés. Or accepterions-nous que nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces soient hébergés dans des hôtels sociaux sans accompagnement ? Accepterions-nous que, à 18 ans, ils soient livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans perspectives, alors même que l'âge moyen de décohabitation se situe, dans notre pays, autour de 25 ans ? Évidemment non ! Alors pourquoi le tolérer pour les enfants qui sont censés être protégés par l'institution ? Comment accepter ces traitements inégaux d'un département à l'autre, ces 101 politiques différentes de protection de l'enfance, qui ne donnent pas aux enfants les mêmes droits selon leur lieu de naissance et de vie Ces situations, qui résonnent comme autant de drames humains, étaient encore méconnues il y a quelques années, mais elles ont fait l'objet de reportages, de témoignages et de mobilisations qui ont permis d'éveiller la société. Grâce à des lanceurs d'alerte, à des travailleurs sociaux dévoués et à d'anciens de l'ASE, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Un seul intérêt doit guider nos débats : celui de l'enfant, supérieur à toute autre considération. C'est pourquoi nous proposerons de revenir au délai d'un an initialement prévu pour la mise en oeuvre de l'interdiction de l'hébergement hôtelier. Cette problématique nous rappelle tristement le drame survenu il y a deux ans, presque jour pour jour. Le 20 décembre 2019, Jess, 17 ans, placé à l'aide sociale à l'enfance, était poignardé à mort dans un hôtel social de Suresnes, ma commune, par un autre enfant placé. Vous aviez d'ailleurs immédiatement réagi, monsieur le secrétaire d'État, en saisissant l'IGAS. Nous devons le dire avec force : en aucun cas, l'hôtel ne constitue un hébergement adéquat pour un enfant. La présence systématique d'un avocat pour les mineurs faisant l'objet d'une procédure d'assistance éducative constitue également un élément essentiel. Garant du secret professionnel, il est en effet un interlocuteur privilégié pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, l'accompagnement des jeunes majeurs sera au coeur de notre débat. Les chiffres, nous les connaissons : un quart des sans domicile fixe (SDF) de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés et 70 % de ces derniers Posons-nous la question : est-il pertinent d'investir autant dans la protection d'un enfant pour que, finalement, le jour de ses 18 ans, tout s'arrête, alors qu'il suffirait de quelques années supplémentaires pour permettre une insertion pleine et entière

chers collègues, ce texte est important, car il est attendu par les travailleurs sociaux, par le secteur associatif et par les enfants eux-mêmes, ainsi que par ceux qui oeuvrent chaque jour pour que ces enfants puissent se reconstruire, mener une vie normale, s'épanouir et s'insérer durablement dans notre pays.

Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance [ ...]. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains.

support de la réforme globale de la protection de l'enfance annoncée de longue date par le Gouvernement et il contient des avancées essentielles, du point de vue tant de la gouvernance que de l'organisation et de l'encadrement. Néanmoins, de nombreux sujets cruciaux pour la protection de l'enfance n'y sont pas abordés : nous attendions particulièrement une réponse aux difficultés d'accès aux pédopsychiatres, un renforcement de l'accompagnement à la parentalité au titre de la prévention, une protection spécifique des enfants vulnérables aux violences numériques et, enfin, un effort de codification législative, au travers de la création d'un code de l'enfance et de la jeunesse. Territoires serait également favorable à la création d'un ministère régalien de l'enfance et de la jeunesse, qui regrouperait les compétences partagées jusqu'à présent entre trois ministères éducation, affaires sociales et justice. Un seul code et un seul ministère permettraient ainsi de mener une politique unifiée. Sur le premier point que j'ai évoqué, la situation est alarmante : nombre d'enfants de l'ASE ne bénéficient pas du suivi d'un pédopsychiatre, alors qu'ils en auraient besoin. Le dernier rapport du Défenseur des droits sur l'accès des enfants à la santé

Monsieur le secrétaire d'État, nous ne pouvons rester passifs face à ce problème. Dans l'attente d'une solution viable, serait-il envisageable de permettre à tous les enfants de l'ASE de bénéficier d'au moins une séance par an chez un psychologue Ce serait également un moyen de détecter rapidement les situations de violence au sein des familles d'accueil ou des foyers, ainsi que les cas fréquents de prostitution. En effet, le rapport, qui vous a été remis le 20 novembre dernier, monsieur le secrétaire d'État, dresse un constat inquiétant à ce sujet. De très jeunes enfants sont concernés, sans avoir conscience de la gravité de la situation. Le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre du premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, le 15 novembre dernier. Jusqu'à 10 000 enfants sont victimes de prostitution en France et les enfants de l'ASE y sont particulièrement exposés. Aussi devons-nous exercer une vigilance toute particulière à leur égard. Le texte comprend des avancées importantes, que nous saluons : l'interdiction du placement à l'hôtel, le contrôle renforcé des professionnels de la protection de l'enfance, la valorisation des assistants familiaux, la rénovation de la gouvernance et l'accompagnement des jeunes issus de l'ASE. Nous sommes également favorables au dispositif de parrainage, dont les contours restent à préciser. De façon complémentaire, à l'aide du levier associatif, il faudrait favoriser le mentorat entre les enfants de l'ASE et les étudiants de grandes écoles, ainsi que l'accès à la culture et aux loisirs, comme le rappelle Gautier Arnaud-Melchiorre, dans le rapport précité. Enfin, nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de la prévention dans le domaine sanitaire et dans le domaine social. Souvenons-nous de la fragilité de l'enfance : comme le disait si bien l'ancien sénateur Michel Amiel : « Un enfant considéré comme normal peut basculer à tout moment et, si un enfant en danger peut devenir dangereux, un enfant dangereux, lui, est toujours en danger. » Ce projet de loi apporte une pierre supplémentaire à l'édifice de la protection des enfants et constitue un rempart contre la violence, un rempart contre la violence, le délaissement et la précarité, que nous ne manquerons pas de consolider en tant que de besoin. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte.

du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Notre pays a toujours porté une attention particulière à la protection des enfants. Dès le XVIII siècle, Jean-Jacques Rousseau rompait avec la conception antique de l'enfance et invitait ses contemporains à considérer l'enfant comme un être à part entière.

je tiens à saluer le travail réalisé par l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance, alors que tous les services de l'ASE ont connu une augmentation importante du nombre d'enfants confiés au cours des dernières années.

Depuis des années, le président du conseil départemental est le chef de file de la protection de l'enfance. Chaque jour, les services départementaux accompagnent des milliers d'enfants placés sur l'ensemble du territoire,

Dans son rapport, notre collègue Bernard Bonne- je salue d'ailleurs la qualité de son travail, fruit de sa parfaite connaissance du sujet en tant qu'ancien président de conseil départemental -parle d'une politique publique qui « manque [ ...] d'efficience

J'approuve également l'élargissement des possibilités d'accompagnement des enfants protégés et l'instauration du parrainage des enfants de l'ASE par des personnes bénévoles. Le parrainage est un mode d'accompagnement

Toutefois, je m'interroge sur les conséquences pratiques de cette mesure. En effet, cela pourrait engendrer une charge supplémentaire importante pour les services des conseils départementaux.

l'une des missions principales est la participation à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance. Nombreux sont les conseils départementaux qui se désolent de son absence à leurs côtés. sans des moyens humains et financiers. Comment pérenniser des revalorisations salariales sur le temps long ? Comment avoir la garantie que les surcoûts engendrés seront bien compensés par l'État ?

après l'abandon du projet de loi relatif à l'autonomie, vanté, cinq ans durant, comme le grand chantier social du quinquennat, le projet de loi relatif à la protection des enfants devait être l'occasion, pour le Gouvernement, de présenter un texte ambitieux sur l'enfance, marquant une nouvelle avancée après les grandes lois de 2007 et de 2016.

inégalités criantes en matière de santé et de formation, précarité résidentielle des anciens enfants placés, nombreuses ruptures dans le parcours de protection, qui sont facteurs de violences institutionnelles, et perte d'attractivité de certains métiers.

l'interdiction du réexamen de la situation d'un MNA ou encore l'augmentation et la sécurisation de la rémunération des assistants familiaux.

Aussi, nous nous opposons au recours obligatoire au fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, ... C'est dommage ! ... perpétuant l'idée du nomadisme des mineurs, phénomène qui n'a jamais été sérieusement documenté. Les bonnes intentions que traduit ce texte restent entachées par ce type de dispositions prises envers les mineurs étrangers, qui ignorent la présomption de minorité et le devoir de protection à leur égard.

Pour permettre aux départements de mettre à l'abri et d'accompagner ces mineurs étrangers isolés, l'État doit soutenir les départements et réduire les différences de charge financière. Un ancien Premier ministre

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires défendra de nombreux amendements en ce sens. Néanmoins, même amendées, les dispositions positives du texte risquent d'être insuffisantes, comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l'homme,

La médiatisation de l'aide sociale à l'enfance a mis en lumière un système trop souvent maltraitant, souffrant des réductions budgétaires des départements et d'un manque de personnel suffisamment formé et reconnu.

Je remercie également l'association Repairs!, Léo Mathey, Lyes Louffok et Juliette Gallouin, de leur expertise. L'amélioration de la coordination entre les acteurs ne suffira pas pour remédier à l'absence de politique globale en faveur de l'enfance et aux conséquences désastreuses de nombreuses mesures mises en oeuvre par différents gouvernements.

La priorité doit être donnée à l'amélioration de la prise en charge des enfants par l'aide sociale et des conditions de travail des assistants familiaux. La prise en charge des enfants concerne évidemment l'accompagnement éducatif en établissement, mais également l'accompagnement médical, y compris en termes de santé mentale.

projet de loi prévoit différentes mesures positives pour améliorer la prise en charge des mineurs de l'ASE. Je pense par exemple à la création d'une base nationale des agréments des assistants familiaux, au renforcement de la place des tiers dignes de confiance, à un meilleur pilotage national, à la non-séparation des fratries ou à l'interdiction des placements à l'hôtel.

Quant aux travailleurs sociaux, qui sont des femmes à 96 % et dont le rôle est primordial pour la protection de l'enfance, ils subissent l'absence de reconnaissance de leur métier et les disparités départementales.

pour l'accueil du premier enfant constitue un progrès qui ne doit pas remettre en cause la majoration pour l'accueil d'un deuxième enfant. Enfin, pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés, ce texte rend obligatoire la présentation des jeunes se déclarant mineurs en préfecture, ainsi que l'utilisation du fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, qui était facultative jusqu'à présent. Cette mesure n'a rien à voir avec la protection de l'enfance, mais relève uniquement du contrôle migratoire. La Défenseure des droits, Claire Hédon, s'est inquiétée, dans son rapport sur ce projet de loi, de l'existence « d'un droit spécifique des MNA, de plus en plus éloigné de la protection de l'enfance Même si des progrès sont accomplis avec ce projet de loi, un écart important reste à combler pour que chaque enfant soit réellement un sujet de droit, pour faire sortir 3 millions d'enfants de la pauvreté et pour consolider et améliorer des services publics réservés à l'enfance, dotés de moyens humains et financiers

C'est une chance, pour eux comme pour nous, que quelques personnes résilientes, hélas trop rares, puissent porter au plus haut niveau de l'État la voix de ces jeunes êtres en souffrance. En effet, 40 % des SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. Parmi ces derniers, 70 % sortent de l'ASE sans diplôme. Ce constat humain est glaçant. le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est bienvenu, même s'il aurait pu être plus ambitieux. Il risque de nous laisser, une fois de plus, dans une forme de frustration.

Actuellement, la première inégalité est sans doute là : situations totalement hétérogènes, politiques et moyens disparates selon les territoires. Je crains que ce texte n'apporte aucune d'avancée en Il faut ensuite donner aux enfants la possibilité de construire une relation affective structurante, que ce soit grâce aux tiers dignes de confiance, qui devraient pouvoir prendre toute leur place lorsque les parents sont défaillants, défaillants, grâce à un dispositif de parrainage ou bien grâce aux frères et soeurs, si on veille impérativement à ne pas séparer les fratries. Votre texte ouvre, sur ces points, des possibilités très intéressantes. Cependant, est-ce suffisant ? Une responsable associative me livrait cette métaphore : « une plante que l'on dépote et rempote sans arrêt ne peut pas s'enraciner. » Il faut impérativement permettre aux enfants de l'ASE de prendre des racines affectives dans des foyers ou auprès d'adultes leur permettant de se construire. Nous connaissons encore tous des exemples d'enfants confiés à des tiers aimants, que l'administration décide de déplacer, dans d'épouvantables déchirements, afin, semble-t-il, d'éviter- on ne sait pourquoi ! -un attachement réciproque. Face à ces situations, il faut veiller à renforcer la formation, tracer une ligne politique claire, permettre les recours, ouvrir aux fonctionnaires la possibilité d'être familles d'accueil.

Comme le disait encore Perrine Goulet, « il nous faut lever les tabous qui traînent depuis si longtemps » et « permettre à chacun de ces oubliés de la République d'avoir un avenir ». La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Je rappelle que, dans notre pays, plus de 300 000 enfants bénéficient chaque année d'une mesure de protection le législateur se doit de suivre, d'améliorer et d'actualiser les mesures visant à garantir un cadre de développement efficace et digne à chaque enfant. Le groupe du RDSE est d'autant plus sensible à cette question que nous avions fait adopter par le Sénat en mai 2020, sur l'initiative de notre ancienne collègue Josiane Costes, une proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement C'est pourquoi je salue l'initiative de ce texte, qui soulève des enjeux primordiaux et introduit de nouveaux outils pertinents et humains, afin de renforcer l'édifice institutionnel relatif à la protection des enfants.

Cette stratégie visant à atténuer les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance est positive, dans la mesure où elle permettra à ces enfants de disposer des moyens de se construire une vie stable. Je rappelle que, aujourd'hui, 70 % des jeunes de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas de diplôme et qu'une personne sans domicile fixe sur quatre vient de la protection de l'enfance. Nous ne pouvons pas tolérer une telle situation.

La Haute Autorité de santé le rappelait déjà en 2017, ces enfants sont plus sujets aux souffrances, inhibitions et troubles psychiques que la population générale.

La situation demeure fragile, malgré la création entre 2018 et 2019 de dix postes d'assistants-chefs de clinique en pédopsychiatrie. Nous attendons un renforcement des actions proposées dans la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie présentée en 2018 par Agnès Buzyn. Je me pose également la question de l'applicabilité effective de la compétence en matière de protection de l'enfance des départements. Nous devons absolument veiller à leur juste association dans le processus d'exécution, au regard de l'aspect financier. Le Gouvernement a déjà débloqué 600 millions d'euros dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous assurer de la soutenabilité financière, pour les départements, des mesures que nous adoptons ? ? Même si ce texte présente quelques failles, le groupe du RDSE le soutiendra, car il apporte des réponses à l'un des enjeux majeurs du XXI siècle, à savoir la protection de l'intérêt de l'enfant.

Quels sont les enjeux d'un nouveau texte sur la protection de l'enfance ?, c'est la seule question qui vaille. Avec ce texte, sommes-nous en mesure de mieux protéger les enfants ? Nous donnons-nous réellement les moyens d'améliorer leur prise en charge ?

Le Gouvernement a-t-il fait le choix de doter la politique de l'ASE de moyens humains et financiers à la hauteur ? La réponse est non ! Les traitements des personnels des établissements de la protection de l'enfance ne sont pas revalorisés ; ils demeurent écartés du Ségur.

Une question demeure essentielle : était-il pertinent de remettre l'ouvrage sur le métier en matière législative ? Nous en sommes à la troisième réforme de la protection de l'enfance depuis quatorze ans. L'État gagnerait à intensifier l'application, l'évaluation et la mise en oeuvre ma collègue Laurence Rossignol reviendra sur ce point. Ce projet de loi tire son origine de la volonté de modifier la gouvernance du secteur, vieux mantra de la DGCS

Renforçons plutôt l'approche partenariale au sein des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. Au fil de l'examen, nous présenterons notre vision de la protection de l'enfance : des établissements et services qui placent le bien-être et la santé globale des enfants protégés au coeur de leur projet et excluent, à l'instar des familles, tout recours aux violences éducatives ordinaires, des services judiciaires qui prêtent attention à l'expression de tous les enfants. En outre, nous pointerons les insuffisances

si la commission des affaires sociales a adopté le projet de loi qui nous est présenté, elle l'a fait après l'avoir modifié par 54 amendements ! Dans notre hémicycle, nombreux sont ceux qui, comme moi, ont siégé au sein de leur conseil départemental. Nous le savons, en matière de protection de l'enfance, les inégalités territoriales sont criantes. Ces inégalités sont d'autant plus inacceptables qu'elles concernent des enfants en réelles difficultés. Les gouvernements ne peuvent plus se satisfaire de belles annonces, qui, une fois les caméras éteintes, ne se traduisent pas concrètement sur le terrain. La politique publique de protection des enfants, si elle est au coeur de nos valeurs républicaines, a un coût. un coût. Parce que ce coût est élevé, nous devons nous assurer de l'efficience de cette politique. Nous le constatons, ses acteurs sont insuffisamment coordonnés. Nous ne pouvons accepter de telles déperditions d'énergie et de moyens.

Si le texte initial étendait les possibilités d'accompagnement en consacrant le parrainage par des personnes bénévoles, notre commission a souhaité favoriser spécifiquement ce dispositif pour les MNA, afin de faciliter leur intégration.

s'agit en effet d'établir rapidement sa situation, afin qu'il puisse, dans le meilleur des cas, entreprendre les démarches auxquelles il peut prétendre. rappelons-le, aujourd'hui, l'accueil de mineurs à l'hôtel ne fait l'objet d'aucun encadrement. Aucun ! L'article 3 de ce projet de loi limite strictement l'accueil dans les hôtels et dans les structures jeunesse et sport aux situations d'urgence, pour deux mois maximum et avec un suivi éducatif. Précisons-le tout de suite, afin que les départements puissent se préparer à cette évolution dans de bonnes conditions, la commission a rendu cette interdiction applicable au bout de deux ans. Pourquoi avons-nous donné plus de temps aux départements ? Parce qu'ils manquent cruellement de moyens, monsieur le secrétaire d'État, alors même que l'arrivée en France de ce jeune public relève non pas de leurs compétences, mais bien de la politique migratoire nationale. dans notre rapport, il conviendrait de transférer à l'État l'exercice et le financement de la compétence de mise à l'abri, mais aussi l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures.

La clef de répartition intégrerait aussi les situations socioéconomiques des départements, ce qui donnerait une bouffée d'air aux plus modestes L'article 14 interdit enfin le réexamen de la minorité et de l'isolement des jeunes reconnus comme MNA et orientés dans un département dans le cadre de la péréquation. La commission a d'ailleurs prévu que cette interdiction concernerait également les jeunes confiés directement par le juge des enfants aux départements. d'importance, l'obligation de transmission mensuelle, par le président du conseil départemental, au préfet des informations portant sur la situation des MNA évalués, ainsi que la généralisation du recours au fichier national d'appui à l'évaluation de la minorité. La commission a approuvé ces obligations, qui permettront d'assurer une péréquation plus juste, en plus de mettre fin au nomadisme administratif, lequel entraîne un grand nombre de doublons. Pour conclure sur le travail mené par la commission, nous avons tenu à préciser que les MNA confiés à des tiers dignes de confiance bénéficient du même régime d'obtention d'un titre de séjour que ceux qui sont confiés à l'ASE.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant d'en venir au fond, je tiens à saluer et à remercier notre collègue Bernard Bonne de la qualité de son rapport, qui éclaire nos travaux. « Quand il s'agit des enfants, la loi ne doit plus être la loi ; elle doit être la mère », disait Victor Hugo, notre illustre prédécesseur. L'intérêt supérieur de l'enfant est la boussole républicaine que le droit pérenne et la loi passagère tentent de suivre. Telle est la règle : qu'il soit un enfant placé, un enfant non accompagné, un enfant isolé ou en danger, un enfant est avant tout un enfant tout court. Ce projet de loi a le mérite de revenir sur les situations difficiles que vivent les mineurs français et étrangers sur notre sol. étend les droits des mineurs et permet de mieux les orienter au sein des dispositifs d'accompagnement de l'aide à l'enfance. Il favorise aussi une meilleure uniformisation de la gouvernance nationale au service des enfants et rappelle l'intérêt du recours au tiers digne de confiance. Toutefois, ce projet de loi aurait pu être plus ambitieux. Il aurait pu mettre en oeuvre les leviers juridiques nécessaires à une protection de l'enfance en général, fondée sur une vision plus intelligente et plus concrète de ce que devrait être la protection des mineurs au XXIsiècle.

Une simple réforme procédurale, associée à des engagements en termes de moyens pour la justice, permettrait de rétablir les déséquilibres et d'orienter davantage les placements vers les tiers dignes de confiance.

les départements, qui ne sont pas toujours à égalité, ont dû gérer l'urgence, tout en essayant de trouver une solution de sortie de ce dispositif. Je me réjouis que l'État trouve une voie de sortie en accord avec les départements. Chaque mineur non accompagné doit pouvoir trouver une solution, adaptée à son âge et conforme à l'objectif de regroupement des fratries. Je conclurai, monsieur le secrétaire d'État, en saluant le travail quotidien des familles d'accueil, des services sociaux à l'enfance, des éducateurs, des animateurs et de tous ceux qui oeuvrent au bien-être de l'enfant.

épuisé, débordé et démoralisé, qu'il s'agisse du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales, qui sont les deux juges importants en matière de protection de l'enfance. Nombre de mes collègues ont évoqué le manque de moyens. Manquer de moyens signifie pour les

De fait, l'urgence est malheureusement caractéristique et symptomatique des situations nécessitant la protection d'un enfant. D'un côté, on prend des précautions dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'autre, on risque de les rendre inapplicables, l'urgence

Le maintien de cette dérogation n'empêchera pas, de toute façon, le juge de confier l'enfant à un tiers en urgence s'il dispose des informations lui permettant de le faire et de considérer qu'il s'agit de la meilleure option dans l'intérêt de l'enfant. Si le juge doit décider en urgence, rien ne l'empêchera ensuite de réviser sa décision, sur la base de l'évaluation des services de l'ASE.

question de les confier à un tiers digne de confiance ou à un membre de leur famille. Le code de procédure civile ne prévoit l'audition de l'enfant que dans le cas où ce dernier est capable de discernement. Pourtant, la notion même de discernement et l'âge à partir duquel l'enfant est considéré comme discernant posent question. Le Syndicat de la magistrature, dans son avis sur le projet de loi, souligne que « les juges des enfants disposent trop souvent d'un temps insuffisant pour les audiences en raison du nombre de dossiers qu'ils ont ce qui les conduit à fixer arbitrairement un âge en deçà duquel ils ne convoquent pas les enfants ». Nous faisons donc face à une contrainte de moyens. Cette situation est dommageable, car, selon le même syndicat- de concert avec toutes les associations -, l'audition d'enfants, même jeunes, présente un réel apport dans la compréhension de la de la dynamique familiale et de la situation de danger. Un enfant, quel que soit son âge, est en mesure d'exprimer- à sa manière, bien sûr -son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l'accueillir.

L'Assemblée nationale a souhaité que le juge des enfants puisse auditionner les enfants capables de discernement. Il s'agit ainsi de replacer l'enfant au coeur de la procédure et de trouver une solution qui corresponde le mieux à ses besoins.

Nous pensons qu'un enfant, quel que soit son âge, est capable d'exprimer à sa manière son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l'accueillir. Dans ces conditions, il ne nous semble pas opportun de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.

un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, alors que l'article 1 ne prévoit qu'une obligation d'entendre le mineur capable de discernement. Nous avons déjà rejeté un amendement

Toutefois, poser une obligation d'entendre l'enfant, même non discernant, dans ces seules situations revient à créer une dérogation peu opportune. En effet, le code civil pose le principe selon lequel l'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge pour toute procédure le concernant. Il ne me ne me semble pas justifié de déroger à ce principe dans ce seul cas particulier. Par ailleurs, cette obligation ne pourra pas être respectée, en pratique, pour des enfants très jeunes qui ne sont pas capables de s'exprimer. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable

vise à prévoir une sanction de caducité si la mesure de placement, lorsqu'elle est prise en urgence et donc sans évaluation préalable, n'est pas suivie des investigations prévues par l'article dans un délai de trois mois.

Le code de procédure civile impose déjà des délais contraignants au juge en matière d'assistance éducative. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, celui-ci les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision. La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires. Puisque l'article 1 impose l'évaluation de l'option chez un tiers avant la décision du juge, cas d'urgence, cette nouvelle obligation s'inscrira dans les contraintes de délais déjà prévues. Poser une nouvelle contrainte de délai n'est donc pas nécessaire et risque de fragiliser juridiquement les décisions du juge des enfants. La commission émet donc un avis défavorable sur cet

le membre de la famille est informé par le juge des enfants de la possibilité de solliciter auprès de lui un accompagnement renforcé, tel qu'une action éducative en milieu ouvert. ouvert. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l'ASE en l'absence de mesure d'AEMO. Cependant, la désignation d'un référent de l'ASE n'est pas, en pratique, de nature à permettre un suivi rapproché du mineur confié, contrairement à une mesure d'AEMO. Faire reposer la mise en place de cette AEMO sur la demande expresse du tiers digne de confiance ou du membre de la famille pourrait constituer un bon compromis et permettre d'augmenter la portée de l'accompagnement offert à ces derniers. La parole

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a proposé que, en l'absence de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance accompagne la personne à qui l'enfant est confié. Pour autant, dans les faits, la désignation d'un référent de l'ASE n'est pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié, contrairement à une mesure d'AEMO.

ou le membre de la famille est informé de son droit à solliciter auprès du juge un accompagnement renforcé, tel qu'une mesure d'AEMO. Cette information nous semble essentielle afin que tous les outils existants soient sollicités, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les personnes visées par l'article 1 puissent être informées de leur droit à désigner soit une personne qualifiée soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elles rencontrent. Quel est l'avis de la commission ? Il est en effet

que toute personne qui bénéficie d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance est informée par les services du département de ses droits et obligations et qu'elle peut être accompagnée dans toutes ses démarches, ce qui comprend donc le droit à bénéficier des mesures visées par les amendements.

le juge des enfants tiendra une audience avec l'ensemble des parties, au cours de laquelle il les informera, conformément à ce qui est prévu dans le code, des différentes possibilités envisagées et des modalités d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Ces amendements étant satisfaits, j'en demande le retrait.

La commission a déjà apporté des précisions dans cet article inséré par l'Assemblée nationale afin de s'assurer de l'effectivité de la mesure. La rédaction que tend à proposer le présent amendement sécurise davantage le dispositif et permettra de bien viser les situations de placement avec résidence de l'enfant à domicile.

Les sommes sont versées sur un compte de dépôt spécialisé et conservées jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants. Le présent amendement tend à prévoir la possibilité, pour le juge, de réserver à l'enfant placé, sur le modèle de ce qui se pratique pour les allocations de rentrée scolaire, tout ou partie des allocations familiales qui sont aujourd'hui versées à l'ASE, sauf décision exceptionnelle du juge. Ce dispositif a vocation à augmenter les moyens de l'enfant en difficulté sociale, dans la perspective de sa majorité ou de son émancipation. Rappelons Rappelons en effet qu'une large part des jeunes sans domicile fixe sont d'anciens enfants confiés à l'ASE, qui ont, la plupart du temps, rompu avec leur famille au sens large. Ce dispositif vise ainsi à enrayer la précarité structurelle des anciens enfants confiés à l'ASE, sur le modèle de la de la réforme des allocations de rentrée scolaire engagée en Actuellement, les allocations familiales dues au titre des enfants accueillis par l'ASE sont reversées au département, dans la mesure où celui-ci assume la charge des enfants qu'il accueille. Le juge peut toutefois décider de les maintenir à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Par ailleurs, depuis la loi de 2016, l'allocation de rentrée scolaire due pour ces enfants est consignée à la Caisse des dépôts et consignations et les sommes accumulées sont reversées à l'enfant lorsque celui-ci atteint sa majorité, afin de l'accompagner dans sa prise d'autonomie. sur le territoire français, de notre ancienne collègue Josiane Costes, la commission a considéré que le droit actuel assurait un équilibre satisfaisant entre versement des allocations au service de l'ASE, avec possibilité de maintien à la famille, et versement de l'allocation de rentrée scolaire à la Caisse des dépôts et

relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge. de loi avait été très largement adoptée par le Sénat le 27 mars 2013, avec les voix de nos collègues socialistes et communistes.

Il vise à renforcer la place des départements dans le processus qui permet au juge de moduler le versement des allocations aux familles qui n'assument pas la charge des enfants. Quel est l'avis de la commission ? Cet

Les travaux de la rapporteure de ce texte pour la commission des affaires sociales, notre collègue Véronique Guillotin, avaient permis de constater que le maintien des allocations à la famille, sur décision du juge, était décidé dans environ la moitié des cas, ce qui permet de relativiser le constat que vous dressez. Par ailleurs, le maintien partiel proposé dans l'amendement aurait une portée limitée. Le juge pourra, par exemple, décider, selon la situation, de maintenir à la famille un montant partiel d'allocations très proche du montant intégral, s'il considère ce maintien justifié. En outre, le fait de fixer dans la loi un plafond de 35 % du montant des allocations pouvant être maintenues à compter du quatrième mois risque de figer un niveau qui ne sera pas forcément adapté. Enfin, une telle mesure pourrait désinciter

quand elle l'est, dans des conditions allégées. Certains départements- les Hautes-Alpes, le Loiret, l'Indre ou les Pyrénées-Atlantiques -n'adressent pas systématiquement de demande de tutelle

entre un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, décidé par le juge des enfants, et le transfert de la tutelle au conseil départemental par le juge des tutelles. Notre amendement vise à corriger ces dysfonctionnements en permettant la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs, aux fins d'ouverture d'une d'ouverture d'une mesure de tutelle. De même, il tend à circonscrire la possibilité d'accomplir des actes non usuels au temps strictement nécessaire à l'ouverture de cette mesure de tutelle, afin de limiter les excès dans l'utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA et de protéger en conséquence les droits et les intérêts de ces enfants. L'amendement

l'amendement n° 57 rectifié . Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, aux fins d'ouverture d'une délégation totale partielle de l'autorité parentale. Cette avancée permettrait notamment de faciliter l'ouverture d'une délégation de l'autorité parentale pour les mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance.

recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ». Cet amendement vise à prévoir que le mineur qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative peut saisir le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Quel est l'avis de la commission ? Les amendements

que le temps nécessaire à l'ouverture d'une tutelle ou d'une délégation plus pérenne de l'autorité parentale. L'intention des auteurs de ces amendements est parfaitement louable. Il s'agit de tirer les conséquences de la trop faible application du code civil, s'agissant de l'ouverture de la tutelle pour les MNA. délimiter ainsi la possibilité d'autoriser la personne accueillant les MNA à réaliser des actes non usuels n'emporte aucun effet utile, puisque rien ne garantit que les MNA feront davantage l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale.

Un membre de la famille, toute personne physique ou morale ayant recueilli l'enfant, ainsi que le ministère public peuvent demander que l'autorité parentale soit déléguée lorsque les conditions sont réunies. Dans le cas où l'enfant est confié à la protection de l'enfance, le service de l'aide sociale à l'enfance apparaît comme le plus à même de demander que lui soit déléguée l'autorité parentale.

privé de l'exercice de l'autorité parentale par le juge pénal ou par le juge aux affaires familiales, ne recouvre automatiquement cette faculté en cas de décès du parent qui l'exerçait seul. Il s'agit de protéger l'enfant au moment du décès ou de la perte de l'autorité parentale du parent qui l'exerçait seul, avant que le juge ne soit saisi, et non de prévoir que le juge puisse être saisi aux fins de confier l'enfant à un tiers, ce que le code civil permet déjà. Il convient donc de rétablir la rédaction prévoyant que si le père ou la mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, le parent restant exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision Cette rédaction permet d'écarter provisoirement le parent défaillant qui s'est vu retirer judiciairement l'exercice de l'autorité parentale, en raison par exemple de son absence, de sa violence, notamment dans le cadre de violences conjugales, ou encore conjugales, ou encore de sa toxicomanie, dans l'attente de la décision du juge aux fins de délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de la personne ou du service qui a accueilli l'enfant. En outre, dès lors que le présent projet de loi prévoit de supprimer la dévolution automatique de l'exercice de l'autorité parentale prévue à l'article 373-1 373-1 du code civil, en cas de décès ou de perte de l'exercice de l'autorité parentale du parent qui l'exerçait seul, il convient en cohérence de supprimer l'alinéa 1 de l'article 373-3 du code civil. Quel est l'avis de

si l'intention est louable, puisque l'amendement vise à éviter qu'un parent défaillant, voire dangereux, qui a été privé de l'exercice de l'autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, ne recouvre ses droits de manière fortuite, lorsque le parent exerçant l'autorité décède brutalement, les conséquences d'une telle disposition peuvent être incertaines en raison de l'ambiguïté des termes et de la systématisation qu'elle introduit. le parent survivant peut n'avoir perdu que certains des attributs de l'autorité parentale. La commission a donc réécrit l'article pour donner plus de liberté au juge aux affaires familiales qui aura été saisi, afin qu'il puisse confier l'enfant à un tiers si son intérêt l'exige, c'est-à-dire à la personne qui a recueilli l'enfant au décès du parent exerçant l'autorité. Avant de se prononcer, le juge pourra apprécier concrètement les circonstances et constater s'il y a encore lieu ou non de priver le parent survivant du premier des attributs de l'autorité parentale, le droit de garde de son enfant. En outre, toutes les dispositions de droit commun de la protection de l'enfant s'appliquent et le juge des enfants, comme le parquet, peut décider en urgence d'une mesure d'assistance éducative. De même, le juge aux affaires familiales peut être saisi en vue de la délégation de l'autorité parentale ou de son retrait. C'est pourquoi je vous propose de ne pas adopter cet amendement visant à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.

l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 du code civil. La commission des affaires sociales a supprimé la mention « à titre exceptionnel ». Cette suppression ne présente aucune plus-value. Confier l'enfant à un tiers ne constitue pas une décision ordinaire. Le seul intérêt de l'enfant ne représente pas une garantie suffisante dès lors que cette notion est floue et à géométrie variable. Les dispositions actuelles ne font pas de l'hypothèse dans laquelle le parent est privé de l'exercice de l'autorité parentale une condition permettant de confier l'enfant à un tiers. Dès lors, il convient de rappeler le caractère exceptionnel de la mesure, afin que des parents qui exercent l'autorité parentale ne puissent se voir retirer leur enfant que lorsque des conditions exceptionnelles le justifient.

lui permettre de confier l'enfant à un tiers si son intérêt l'exige, et ce afin d'éviter qu'un parent défaillant ne retrouve la garde de son enfant à la mort du parent qui exerçait seul l'autorité parentale.

cet amendement ne présente aucun lien avec l'assistance éducative ou l'aide sociale à l'enfance ». Or ce texte porte non pas sur l'assistance éducative ou l'aide sociale à l'enfance, mais sur la protection des enfants

Ces amendements, souvent identiques ou proches, portaient principalement sur deux thématiques : l'exercice de l'autorité parentale et les violences conjugales. Pour ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale, seul l'article 2 figurait dans le texte initial. Cet article concerne les délégations de l'autorité parentale nécessaires à l'accomplissement des actes par le service gardien de l'enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Par conséquent, les amendements relatifs aux modalités d'exercice et de délégation de l'autorité parentale concernant un enfant faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance ou d'assistance éducative sont compris dans le périmètre le périmètre indicatif du texte adopté par notre commission le 20 octobre dernier. En revanche, sont exclus de ce périmètre les amendements portant sur les conditions de délégation et d'exercice de l'autorité parentale sur tous les enfants, sans condition. condition. Aucune disposition du texte déposé ne porte par ailleurs sur la prévention et la lutte contre les violences conjugales, ni sur les effets de ces violences sur les mineurs qui y sont exposés. C'est pourquoi la commission a considéré que des amendements portant sur de telles dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi. projet de loi. Celles-ci figuraient en revanche au coeur des textes que nous avons examinés récemment, comme la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié,

est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à préciser que l'intérêt des frères et soeurs de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative doit être pris en compte au même titre que celui de l'enfant lui-même avant d'envisager un accueil de la fratrie. Cette précision est en réalité satisfaite par le présent article. Un enfant est confié avec sa fratrie à un établissement ou à une personne seulement si ses frères et soeurs font eux-mêmes l'objet d'une mesure éducative. L'article, qui prévoit que l'enfant est accueilli avec ses frères et soeurs sauf si son intérêt commande une autre solution, s'applique donc à chacun d'entre eux. Le juge prendra en compte l'intérêt de chaque enfant de la fratrie avant de se prononcer. La commission émet donc un avis défavorable

En effet, quand un enfant exprime le souhait de ne pas être remis en contact avec l'un de ses parents, ou les deux, il faut qu'il puisse être entendu. Quel est l'avis de la commission ? Nous sommes tout à

durant la durée d'une ordonnance de protection. Or M. le rapporteur a expliqué que les dispositifs votés en 2019 et 2020 étaient trop récents pour être évalués et pour modifier le cadre juridique existant. Pour notre part, nous avions déjà souligné que le dispositif proposé en matière d'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales n'était pas suffisant. Nous considérons qu'un conjoint violent ne peut pas être un bon père- cette idée commence d'ailleurs à être partagée.

Parce qu'il s'agit d'un projet de loi sur la protection de l'enfance et parce que les textes actuels ne sont pas suffisants, nous vous proposons de rétablir l'article 2. Nous

les arguments évoqués en commission. Tout d'abord, le régime juridique de l'ordonnance de protection a été modifié par deux lois récentes, en 2019 puis en 2020, afin de faciliter l'accès au juge et de renforcer les mesures de protection des victimes. Il conviendrait donc de stabiliser ce cadre pour qu'il se déploie avant de modifier de nouveau les règles. Ensuite, nous avons considéré que la loi permettait déjà au juge de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Résultat : ces jeunes, en souffrance extrême, peuvent devenir violents les uns envers les autres, comme l'illustre le drame de Jess, un adolescent de 17 ans poignardé à mort par un autre jeune dans un hôtel à Suresnes. Ces mineurs sont aussi la proie de différents trafics, nous le savons.

éléments sur la position à la fois exigeante et pragmatique de la commission. Aujourd'hui, la loi n'interdit pas l'accueil à l'hôtel. On estime qu'environ 7 500 à 10 000 mineurs suivis par l'aide sociale à l'enfance y sont logés. Ce sont en majorité des mineurs non accompagnés.

Merci

des personnes handicapées a rendu une décision d'orientation vers un établissement spécialisé et adapté, qui doit les prendre en charge de manière effective ». Malheureusement,

Dans ce sens,

Quel est l'avis de la commission ? Alors que l'interdiction de l'hôtel et l'encadrement de l'accueil en structures seront applicables au bout de deux ans, il est proposé, avant cette date d'application, qu'un décret puisse fixer pour ce type d'accueil des conditions d'encadrement des mineurs.